La séance est reprise. Nous reprenons l'examen du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

de la commission des lois. Pour faciliter le déroulement des travaux du Sénat, compte tenu des souhaits qui ont été formulés par Mme la présidente de la commission des affaires sociales et par le Gouvernement, je soumets au Sénat deux modifications dans l'organisation de nos travaux.

d'une part, d'une demande de priorité sur les articles 57, 57 et 78 afin qu'ils soient examinés après l'article 38, d'autre part, d'une demande de réserve du chapitre I du titre VII, c'est-à-dire des articles 50 à 52, ainsi que des amendements tendant à insérer des articles qui leur sont rattachés, afin qu'il soit examiné après le chapitre III du titre VII, soit après l'amendement n° 1077 tendant à insérer un article additionnel après l'article 59 Selon l'article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité et la réserve sont de droit quand elles sont demandées par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande La priorité et la réserve sont ordonnées.

Cet amendement vise à étendre la dérogation à l'obligation d'autofinancement aux opérations en investissement réalisées par les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux,

Il autorise les préfets de département à accorder une dérogation à la règle qui impose une participation financière minimale au maître d'ouvrage appartenant au bloc communal- commune, EPCI ou syndicat mixte fermé.

qui ne bénéficient par ailleurs ni d'une fiscalité propre, ni d'un transfert de moyens de la part des collectivités membres, ni de dotations de l'État telles que la dotation globale de fonctionnement (DGF) ou la dotation globale d'équipement (DGE). permettre aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux de bénéficier des mêmes mesures dérogatoires pour conduire les actions environnementales d'intérêt général que les établissements publics des parcs nationaux ou les associations gestionnaires d'espaces naturels.

La plupart des établissements publics en charge de politiques environnementales- parcs nationaux, établissements publics territoriaux de bassin, parcs naturels marins, par exemple -, ainsi que les syndicats mixtes des parcs naturels régionaux sont encouragés à mettre en place une gouvernance ouverte, rassemblant notamment des associations de représentants de la société civile, des organismes socioprofessionnels et des chambres consulaires dans leurs instances de pilotage. En conséquence, le syndicat mixte ouvert dit « élargi » est l'unique structure autorisée par les dispositions législatives actuelles pour la gestion des parcs naturels régionaux. Or une grande majorité d'entre eux sont actuellement gérés par des syndicats mixtes ouverts « restreints car les syndicats mixtes ouverts « élargis » sont exclus du dispositif d'accès au FCTVA, alors même que les organisations socioprofessionnelles ont une part marginale dans le financement et la gouvernance à dominante publique. Cette interdiction constitue un frein financier majeur à la mise en place d'une gouvernance ouverte sur le territoire des parcs. Il est donc proposé d'y remédier.

et n'a pas vocation à évoluer, car l'objectif du FCTVA est toujours resté le même : soutenir l'investissement des collectivités locales et de leurs groupements. Ainsi, les groupements de collectivités locales sont éligibles au FCTVA seulement

au-delà des seuls syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux. Cela ne manquerait pas, à terme, de susciter de nouvelles demandes d'élargissement du champ des bénéficiaires. Au demeurant, l'enveloppe du FCTVA vient déjà d'augmenter cette année, sous l'effet de l'automatisation de la procédure.

lors des procédures d'évaluation environnementale et d'autorisation environnementale. Les 56 parcs naturels régionaux couvrent à ce jour 17,5 % du territoire national et constituent des territoires très majoritairement ruraux. Les projets y sont par conséquent peu nombreux, mais leurs impacts au regard des critères de classement peuvent être importants. Rétablir une consultation obligatoire des parcs naturels régionaux dans le cadre de certaines procédures

Les différentes réformes liées aux autorisations environnementales ont grandement fragilisé le cadre de concertation qui permettait jusqu'alors aux parcs naturels régionaux d'assumer leurs obligations en matière de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire. Les situations qui entourent la réalisation de projets nécessitant une évaluation environnementale ou une autorisation sont aujourd'hui floues et soumises à des appréciations locales sans réelle cohérence d'un territoire à l'autre.

d'ailleurs, nous avons un partenariat avec eux dans le cadre de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ils accompagnent ainsi nos territoires en amont. C'est, je crois, beaucoup plus efficace que de multiplier les procédures formelles. Il n'est donc pas souhaitable de revenir sur les récentes

Il vise une application du principe de différenciation sur ces territoires et offre aux parcs naturels régionaux la possibilité, dans le cadre de la réglementation existante et sous contrôle du préfet, de procéder à une adaptation des seuils de déclaration et d'autorisation administrative requises en application du code de l'environnement et du code forestier. Cette disposition permet une plus grande prise en compte de la sensibilité de tout ou partie des territoires d'un parc. En effet, chaque parc naturel régional est doté d'une charte et d'un plan qui fixent les orientations d'aménagement et de protection du territoire. Les enjeux paysagers et de biodiversité y sont identifiés et des objectifs de préservation sont fixés. Si la charte ne réglemente pas les activités qui se déroulent sur le territoire, elle a pour vocation de garantir leur compatibilité avec les objectifs de protection. La légitimité des parcs en la matière repose également sur leur gouvernance mixte. L'État est cosignataire de la charte et classe le territoire par décret. Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional est administré par un organe de gouvernance réunissant l'ensemble des collectivités territoriales : communes, intercommunalités, régions et départements. Il a pour responsabilité de mener la concertation locale en y associant les parties prenantes, notamment les chambres consulaires. Par une mise en oeuvre du principe de différenciation à l'échelle des parcs naturels régionaux, il est proposé de mieux répondre à l'attente des élus locaux et des citoyens et de rendre plus efficace l'action des parcs dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie des aires protégées. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone,

Ils voient leurs administrés se calfeutrer chez eux en période d'épandage ; ils voient les taux de contamination des riverains dépasser les seuils autorisés ; ils doivent prendre des décisions pour le bien commun,

le pire, plus de 120 municipalités ont ainsi pris des dispositions de protection des habitants résidant à proximité des lieux d'épandage. Le temps de nos concitoyens, le temps de la biodiversité n'est pas celui, étirable à l'infini, des lobbies

M. Didier Marie. Cet amendement vise à donner aux maires les outils nécessaires pour garantir le bon entretien des chantiers, lesquels peuvent constituer des foyers importants de désagréments pour les riverains et de nuisances pour l'environnement. le maire soit habilité à édicter des recommandations de bonnes pratiques à destination des parties prenantes, afin d'accompagner le respect par ces dernières des exigences en matière de propreté des emprises de chantier et de préciser le contrôle effectué. effectué. Les sanctions pénales existantes sont, d'une part, insuffisamment dissuasives dans un contexte de multiplication des incivilités et, d'autre part, inapplicables en raison du principe d'imputabilité stricte des infractions pénales. Par ailleurs, alors que la jurisprudence relative au champ d'application matériel des dispositions du code de l'environnement en matière de déchets n'est pas certaine, le présent amendement tend à établir, sans ambiguïté, que le maire peut faire usage de la procédure administrative

? Nos collègues souhaitent, par leur amendement, renforcer les pouvoirs du maire pour garantir le bon fonctionnement des chantiers, lesquels peuvent créer des nuisances pour les riverains et l'environnement.

totalement dépourvue de portée normative. Cela rejoint les discussions que nous avions hier : la loi n'a pas vocation à tout définir ni à tout écrire.

puisque la salubrité publique est l'une des composantes du pouvoir de police générale du maire, qui l'autorise justement à prévenir et à faire cesser les pollutions de toute nature.

attaque contre Mme Hidalgo, qui n'est pas capable de gérer les chantiers de la ville de Paris sans multiplier les zones de turbulences,

que le choix des modalités de collecte et de traitement des déchets par le nouvel EPCI soit fait dans le respect du principe de non-régression, tel que défini à l'article L. 110-1 du code l'environnement.

! Les collectivités territoriales peuvent s'appuyer sur un établissement public territorial de bassin

laquelle est en vigueur pour douze mois encore. Or aux termes de l'article 38 de la Constitution, il n'appartient pas à un parlementaire d'étendre le champ d'une habilitation à légiférer par ordonnances. Dès lors, ces amendements étant contraires à l'article 38 de la Constitution, ils doivent être déclarés irrecevables.

commission des affaires économiques ? Aujourd'hui, rien n'empêche les villes de Paris, Lyon et Marseille de se fixer elles-mêmes des objectifs par secteur géographique. Il me semble que la loi ne résoudrait en rien les difficultés rencontrées dans certaines zones où le foncier est particulièrement rare

En effet, les chiffres de la construction sont au rouge depuis de nombreux mois. On accusera sans doute les maires de ne pas porter l'effort nécessaire en période électorale ou on évoquera les conséquences du covid-19 ... Mais les freins, et donc les leviers, sont plutôt à chercher du côté du désengagement de l'État de l'exercice de ses missions au service du droit au logement pour toutes et tous. Ainsi, si quelques efforts ont été réalisés dans le cadre du plan de relance

l'État doit aussi jouer son rôle, apporter les subsides nécessaires, arrêter de ponctionner le secteur HLM et cesser de faire des économies de bouts de chandelle sur les bénéficiaires

la politique du Gouvernement aura déstabilisé et fragilisé tout un secteur des ponctions de plusieurs milliards d'euros et des réorganisations à marche forcée et sans cohérence, qui éloignent les prises de décision de la réalité des territoires et des attentes des Français.

le problème numéro un de la construction de logements abordables. La dynamique pour réaliser 150 000 logements sociaux par an et libérer des terrains a été brisée dès 2017. entraîné toutes les conséquences que l'on connaît aujourd'hui, au détriment des familles qui n'arrivent pas, avec leurs ressources, à se loger dignement. Aussi ferons-nous des propositions visant à adapter les politiques d'habitat à la diversité des territoires, à en renforcer le pilotage territorial et à donner des outils aux élus pour encadrer le prix du foncier, notamment dans les zones les plus tendues.

pour dégager un maximum de collectivités de leurs obligations en matière de mixité sociale. Je préfère être claire tout de suite : nous voterons contre tous les amendements qui visent à affaiblir, sans raison, la portée de la loi SRU. Nous souhaitons qu'un bilan puisse être réalisé à l'issue de ces débats, après l'application de ce texte, sur les conséquences concrètes de l'élargissement des critères d'appréciation de la pertinence de l'exemption au titre de la mauvaise connexion au bassin de vie et d'emploi, en ne se référant plus à la notion de mauvaise desserte

des contradictions urbaines, notamment lorsque se trouve constatée une densité déjà forte, qui se traduit par des coûts fonciers et des difficultés de libération d'emprises. Par conséquent, l'effort exigé de communes qui se

En quelque sorte- et c'est le point sur lequel il va falloir travailler -, il prévoit une substitution des barèmes et des pourcentages fixés par un système de contrats individualisés. Les autres articles restent en vigueur,

l'horizon, c'est l'augmentation du déficit de logements sociaux, en raison notamment de l'arrêt temporaire des chantiers pendant cette période : on a constaté une baisse de 30 % de la construction de logements sociaux en 2020.

champ d'application de l'article 55 de la loi SRU, qui oblige les communes les plus importantes à disposer d'un taux minimum de logements sociaux par rapport à l'ensemble des résidences principales, les communes nouvelles dont les communes d'origine ne sont pas soumises à cette obligation.

de faire partie d'une agglomération de plus de 30 000 habitants pour être exempté du critère de faible tension sur la demande de logement social. Un certain

l'avis du Gouvernement ? Le seuil de 3 500 habitants, applicable depuis l'an 2000, est aujourd'hui une référence bien connue de tous les acteurs concernés.

dispositifs spécifiques pour les nouveaux entrants, déduction de prélèvements, etc. Ces mécanismes sont d'ailleurs complétés par le présent texte, qui procède à une adaptation substantielle des objectifs de rattrapage triennaux. En conséquence, j'émets à mon tour un avis défavorable.

déficitaires bénéficiant de la DSU sont d'ores et déjà exemptées du prélèvement SRU si elles comptent un minimum de 15 % ou 20 % de logements sociaux.

cet outil permettra de territorialiser les objectifs et de répondre aux desiderata de notre collègue. Aussi, je ne voterai pas ces amendements, malgré toute l'affection que nous portons à Philippe Dallier.

dans un cadre où chacun exerce pleinement ses responsabilités.

fragiliser le nécessaire dialogue avec les communes. Cette possibilité d'appel au préfet à titre gracieux permettra justement d'éviter que les seules issues pour la commune ne soient, de fait, le tribunal administratif

En l'état actuel du droit, ce sont les intercommunalités qui ont le pouvoir de proposer l'exemption de certaines communes de leurs obligations au titre de la loi SRU, elles sont les chefs de file reconnus des politiques locales de l'habitat menées sur les territoires, à travers le PLH. Il est donc tout à fait légitime et cohérent qu'elles constituent le premier échelon de proposition des communes afin que l'exemption potentielle, si elle est accordée par l'État après avis de la commission, puisse être prononcée

En effet, l'objet du projet de loi est, rappelons-le, d'abandonner le critère de faible desserte par les transports en commun, jugé désuet, au profit d'un critère multifactoriel d'isolement. Il s'agit d'une avancée dans les critères d'exemption. Par ailleurs, les communes risquant de ne pas être prises en compte par ce critère le seront par le second, qui porte sur la faible demande

pourtant que la situation des communes rurales ou périurbaines au regard des exemptions sera très sensiblement modifiée, puisque le critère de faible desserte en transports en commun est remplacé par un critère

des affaires économiques ? Monsieur Richard, il me semble que cet amendement est partiellement satisfait. Je vais essayer de vous en convaincre. Vous proposez d'adapter les obligations des communes en fonction du taux d'inconstructibilité sur leur territoire et vous pointez l'effet de seuil

Dans ce texte, nous avons cherché à assouplir les trajectoires et à permettre une meilleure contractualisation afin de prendre en compte les difficultés, mais je ne suis pas favorable à la proratisation sur la fraction du territoire constructible.

Nous sommes bien entendu favorables à la prise en compte des spécificités territoriales, comme l'inconstructibilité ou le recul du trait de côte ; cela contribue à l'adaptation du dispositif SRU aux réalités des territoires et à ne pas aggraver la vulnérabilité Toutefois, l'application des exemptions SRU doit être corrélée avec d'autres restrictions en matière de construction de logements privés ou de locaux d'activités. C'est la raison pour laquelle il ne nous paraît pas opportun de rendre automatique les critères d'exemption SRU plutôt que d'examiner les situations locales en lien avec l'EPCI, comme c'est le cas actuellement.

la non-automaticité de l'exception pour inconstructibilité suscite l'incompréhension des élus et des populations, dès lors qu'il s'agit

de l'amendement n° 1540 rectifié, la commission a émis un avis défavorable, car son adoption conduirait à faire sortir de la loi un très grand nombre de communes, sans que cela soit justifié et sans tenir compte de la nécessité de continuer à construire des logements sociaux

des établissements où les résidents purgent de longues peines. Cet amendement vise par conséquent à ajouter à la liste des logements locatifs sociaux les maisons centrales et les centres de détention.

Catherine Procaccia. Cet amendement a pour objet de permettre le décompte, au titre des logements locatifs sociaux, d'un certain nombre de dispositifs tels que les résidences hôtelières à vocation sociale, qui peuvent accueillir jusqu'à 80 % de personnes en situation de précarité, à la condition que l'occupation de ces logements ou hébergements soit établie depuis au moins un an. Il tend également à permettre le décompte, au titre des logements locatifs sociaux, des hébergements d'urgence recevant des personnes sans abri,

Drexler. Cet amendement tend à comptabiliser les emplacements des aires permanentes d'accueil des gens du voyage dans les quotas de logements sociaux auxquels sont soumises certaines communes. Une telle disposition a déjà été adoptée à plusieurs reprises par le Sénat, sans qu'elle ait été pour autant retenue dans les textes définitivement adoptés. Les aires d'accueil ont pourtant un coût non négligeable pour la collectivité et entrent parfaitement dans le champ des hébergements sociaux. Leur prise en compte dans les quotas SRU permettrait ainsi de reconnaître les efforts fournis par les communes et les EPCI en matière d'accueil des gens du voyage et les inciterait à les poursuivre dans le cadre des schémas départementaux.

sincèrement, si Prévert était encore vivant, il en ferait un inventaire poétique et si Boris Vian était encore vivant, il en ferait une complainte

quels sont ses buts, à quoi il sert, avant de considérer que tous les établissements qui accueillent des enfants de gens qui sont dans les logements sociaux sont eux-mêmes des logements sociaux, que toutes les aires d'accueil pour les gens du voyage sont des logements sociaux, que toutes les casernes militaires sont des logements sociaux. Et pourquoi pas les niches des chiens ?

après la vente des logements locatifs sociaux. Les zones tendues manquent cruellement de logements abordables adaptés aux ressources et aux besoins des Français. Or la durée de dix ans, retenue dans le cadre de la loi ÉLAN n'incite pas les communes à reconstituer rapidement une offre locative sociale. Par ailleurs, dans les territoires en forte tension, il y a un risque de revente avant le délai de dix ans avec une plus-value. Une durée de dix ans est donc trop longue pour garantir une occupation sociale du logement. Notre amendement vise à revenir à une durée de cinq ans pour maintenir une dynamique de production de logements sociaux.

dans les objectifs de réalisation fixés par la loi SRU. Les logements en caserne de la gendarmerie nationale ne peuvent être considérés comme des logements locatifs sociaux. Les inclure dans le décompte des objectifs de réalisations fixés par la loi SRU constituerait- c'est un euphémisme -un affaiblissement de la construction de logements sociaux. Cet amendement vise donc à supprimer ce dispositif. L'amendement n° 1390, présenté Mme la ministre déléguée. Dans le droit fil de ce qui a été évoqué, le Gouvernement propose de revenir sur le retrait de l'inventaire des résidences principales des logements des casernes des militaires de la gendarmerie nationale. En effet, bien que ces logements soient évidemment nécessaires, ce ne sont pas des logements sociaux.

en application de l'article L. 302-5 du code de la construction. Ce serait en effet cohérent avec la politique d'accession sociale à la propriété et de lutte contre l'insalubrité, menée par l'État dans les départements d'outre-mer. Cela représente aussi une nécessité pour nos territoires qui comptent un grand nombre d'habitats indignes et insalubres. Ces logements sont destinés à des ménages aux revenus très modestes et sont un moyen de répondre à la crise du logement outre-mer, dont l'ampleur est autrement plus importante que sur le territoire hexagonal. Cela correspond, enfin, à l'aspiration profonde de nos populations de posséder leur propre logement. En les intégrant dans le décompte, cet amendement vise à encourager leur production par les collectivités ultramarines. L'amendement

? Ces deux amendements reprennent une proposition du rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). Ces logements évolutifs sociaux, que vous souhaiteriez voir entrer dans le décompte des logements au titre de l'article 55 de la loi SRU, sont des logements en accession et amélioration très sociale. Ils visent à lutter contre l'habitat indigne, qui est une réelle source de préoccupation et de difficultés dans les départements et collectivités d'outre-mer. Le rapport note que le fait qu'ils ne soient pas décomptés parmi les logements SRU nuit à leur développement et considère que ces dispositifs sont destinés au même public que les logements locatifs très sociaux. Ce décompte apparaîtrait, toujours selon le rapport, comme pouvant être cohérent avec, par exemple, la comptabilisation des logements en accession sociale à la propriété, introduite

Je note, enfin, que la délégation sénatoriale aux outre-mer n'a pas souhaité reprendre cette proposition dans le rapport qu'elle a établi sur le logement. Par conséquent, la

Un délai de dix ans semble plus approprié, afin de mieux étaler dans le temps les efforts de construction de logements et l'atteinte du taux cible de 25 %. Sortir trop rapidement de ces typologies revient à pénaliser les communes, alors même qu'elles engagent une politique de mixité sociale.

Même avis. Il me semble que la loi ÉLAN a trouvé un équilibre. Par ailleurs, passé le délai de cinq ans, la condition d'occupation sociale n'est plus totalement garantie puisque, en cas de changement de propriétaire, il n'est pas certain que les nouveaux occupants répondent aux critères de plafond de ressources définis par la réglementation. Madame Procaccia, l'amendement

est à Mme Sabine Drexler. L'État doit affirmer sa connaissance des réalités locales et, le cas échéant, acter officiellement les difficultés locales qui freinent les maires volontaires lors des plans triennaux en notant que la période de trois ans est bien trop courte au regard de la complexification de la législation. Une période de cinq ans devrait permettre d'obtenir un bilan plus objectif de la situation. Cet amendement vise ainsi à allonger de deux ans cette période de notification à la commune de l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux en passant d'une période triennale à une période quinquennale.

la vie économique s'est arrêtée, tout comme la construction de logements sociaux. En conséquence, il semble injuste que les communes qui doivent remplir leurs obligations au titre de l'article 55 de la loi SRU soient pénalisées par la non-atteinte des objectifs qui leur ont été fixés. C'est pourquoi cet amendement a pour objet de créer deux « années blanches » pour 2020 et 2021 en termes d'objectifs de construction de logements locatifs sociaux. La période triennale qui a tout juste débuté en 2020 trouvera ainsi son achèvement à la fin de l'année 2024 et non à la fin de 2022.

d'avantages. Je tiens à vous signaler que cela serait de nature à allonger d'autant la durée des pénalités liées, par exemple, au constat de carence ou des prélèvements liés au déficit, alors que la période triennale est, de fait, plus courte. Cette dernière permet de faire deux bilans par mandature et de pouvoir réajuster les choses si, dans le courant du bilan triennal, des efforts ont été faits. De ce fait, les prélèvements, voire les pénalités,

Afin de permettre une meilleure articulation entre la loi SRU et la loi de protection des sites patrimoniaux remarquables (SPR), l'amendement vise à ce que, dans les communes dont une partie du territoire est classée en SPR, la loi SRU ne s'applique qu'à la partie qui n'est pas incluse dans le SPR. En effet, seules les parties non couvertes par le SPR sont soumises au droit commun de l'urbanisme, ce qui justifie que s'y appliquent les mêmes objectifs que dans les autres communes. En revanche, dans la mesure où les parties couvertes par le SPR subissent des contraintes d'urbanisme fortes, elles ne devraient pas être soumises à un objectif de construction tel que celui de la loi SRU. Comme aucune commune ne voit 100 % de son territoire couvert par un SPR, cela n'exempte aucune commune de l'application de la loi SRU. L'objectif de construction de 25 % de logements sociaux entre en contradiction avec le classement de certaines communes en site patrimonial remarquable en vertu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à à l'architecture et au patrimoine. Alors que cette loi vise à protéger des sites présentant un intérêt public du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, elle n'ouvre droit à présent à aucune adaptation de l'objectif de construction de logements sociaux. en résulte différents types de problèmes comme l'absence de foncier disponible, du fait des contraintes d'urbanisme résultant du statut de SPR et des restrictions des possibilités architecturales liées à la hauteur des bâtiments, mais aussi des atteintes à l'environnement du fait de la destruction d'espaces boisés protégés. Il existe actuellement environ 800 sites patrimoniaux remarquables. La parole

Ces deux amendements visent à concilier les obligations issues de la loi SRU et celles qui résultent des sites classés patrimoine remarquable. Leurs auteurs proposent que la loi SRU ne s'applique qu'à la partie non classée du territoire de ces communes. S'il me semble légitime d'articuler les différentes obligations légales s'imposant aux communes, soit en aménageant les objectifs de la loi lorsque c'est indispensable, ce n'est pas certain en l'espèce, soit en aménageant le rythme de rattrapage dans les contrats de mixité sociale dans les autres cas.

Gourault ! Je pense que nous serons en capacité de produire un texte satisfaisant à l'issue de la navette. Toutefois, il reste quelques points sur lesquels le Gouvernement n'est pas d'accord avec la commission, ce qui nous amène à déposer quelques amendements, mais pas énormément. Celui-ci en fait partie.

Aussi, le Gouvernement propose de rétablir les modalités actuelles de décompte en supprimant la pondération des logements en fonction de leur typologie de financement. Il s'agit là d'un des points de dissensus de fond que nous avons avec la rapporteure et la commission. Quel est l'avis de la commission des affaires

nous a montré que, si la loi SRU a effectivement permis d'augmenter la construction de logements sociaux et de mieux les répartir sur l'ensemble du territoire national, il y a un point sur lequel elle n'a pas atteint ses objectifs, c'est celui de la mixité sociale.

très sociaux peuvent avoir besoin d'un accompagnement social renforcé, lequel aura des conséquences pour le budget de la commune, en particulier au niveau

SRU sont incitées à ne construire que des studios ou des logements pour étudiants qui seront comptabilisés dans le quota SRU. Cette politique du logement ne permet pas d'accueillir

que leur nombre parmi les résidences principales. Dès lors, vous l'avez dit également, les maires qui souhaitent faire du chiffre et minimiser l'impact sociologique de la loi SRU sur leur commune ont plutôt intérêt à construire des logements de petite surface destinés aux populations les moins défavorisées,

Grégoire Fauconnier. Celui-ci a montré, dans sa thèse, qu'il y avait effectivement des contournements de la loi SRU, car certaines communes remplissent leurs obligations uniquement par la construction de logements ou de structures pour étudiants ou personnes âgées. De fait, la mixité sociale ne progresse pas. Nous avons également constaté que